disposition va dans le sens du plan Climat du Gouvernement qui vise à éradiquer les passoires thermiques en 2025. Il s'agit non pas de sortir des logements du parc locatif, mais bien d'inciter les propriétaires à faire les travaux.

en kilowattheure d'énergie primaire par an suppose de pouvoir le mesurer avec fiabilité. Or à ce jour le diagnostic de performance énergétique n'est pas fiable.

: La parole est à Mme Nelly Tocqueville. Cet amendement vise une nouvelle fois à structurer les contours du service public de la performance énergétique de l'habitat en apportant aux citoyens une information neutre sur la rénovation énergétique. En effet, une très grande partie des ménages qui font des travaux d'économie d'énergie ne passent pas par ce service public, mais sont contactés par des professionnels qui vendent des certificats d'économies d'énergie,

la libre capacité des entreprises à proposer des offres commerciales aux consommateurs.

le rester pourront le signaler dans un délai de deux ans. Le présent amendement a ensuite pour objet de définir les conditions de transfert ultérieur au réseau public des colonnes montantes dont les copropriétés auront choisi de demeurer propriétaires. Il vise enfin à assurer un règlement pérenne du sujet en intégrant automatiquement toutes les nouvelles colonnes montantes au réseau public.

un transfert possible sur demande du propriétaire dès l'entrée en vigueur de la loi ou, à défaut d'une telle décision, et comme prévu dans l'amendement du Gouvernement, un transfert général de l'ensemble des colonnes à l'issue d'un délai de deux ans, avec possibilité de revendiquer la propriété dans ce même laps Cette alternative permettra notamment aux bailleurs sociaux ou aux copropriétés qui feraient ce choix lors d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de transférer sans attendre leurs colonnes. Pour le reste, le présent sous-amendement vise à apporter plusieurs précisions rédactionnelles et à lever une ambiguïté éventuelle sur un point qui tient à l'obligation de remise des colonnes en bon état de fonctionnement. Celle-ci ne pourra être exigée que des colonnes dont les propriétaires auraient revendiqué et obtenu la propriété dans les deux ans, mais dont ils décideraient par la suite de se séparer. Il s'agit d'un cas très théorique, mais qu'il est nécessaire de prévoir. En revanche, le transfert avant deux ans ou au plus tard

est à Mme Christine Bonfanti-Dossat. Un flou juridique existe quant à la propriété des colonnes montantes d'électricité dans les immeubles d'habitation. Ce fait est particulièrement problématique au regard des coûts importants de rénovation qui sont supportés soit par le distributeur d'énergie, soit par la copropriété. Le 18 janvier dernier, le Gouvernement a émis des propositions, notamment pour recenser les situations et clarifier le statut des colonnes montantes. Or le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique n'évoque pas ce sujet. Cet amendement d'appel vise donc à interroger le Gouvernement sur le calendrier et les moyens qu'il prévoit de déployer, mais comme M. le secrétaire

afin de repositionner le présent article dans la partie du code de la construction et de l'habitation relative à la réglementation sur les bâtiments neufs en y créant un article nouveau. Il tend ensuite à mettre en cohérence cette mesure avec les dispositifs existants dans un souci de simplicité administrative pour les entreprises.

à favoriser l'intérêt général en matière de transition énergétique et, enfin, à conforter pleinement le lien apporté par la construction biosourcée dans la cohésion des territoires et la solidarité entre L'article 55 B nouveau du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique complète et précise les dispositions relatives à la performance énergétique et environnementale des bâtiments du code de la construction et de l'habitation telles qu'issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, et de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dont le VI de l'article 14 dispose : « L'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. En précisant que la déclaration environnementale de performance des produits de construction devra faire mention, parmi d'autres critères, de la quantité de matériaux biosourcés qui seront incorporés, l'article 55 B, dans sa rédaction initiale, relevait donc d'un motif d'intérêt général prédéfini par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il convient de maintenir l'incitation explicite en faveur des matériaux biosourcés, afin de donner toute son efficacité à la future loi.

à partir du 1 janvier 2020. Cet amendement tend à rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale, qui a introduit l'opposabilité du diagnostic de performance énergétique. Cette mesure nous semble fondamentale dans le cadre de nos efforts pour lutter contre la précarité énergétique et contre le gaspillage d'énergie. Aujourd'hui, le DPE n'est pas obligatoire,

Le rendre opposable permettra de responsabiliser tous les acteurs et de fiabiliser les DPE. Par ailleurs, la commission a motivé la suppression du présent article par le manque de fiabilité des DPE.

et le ministre de la cohésion des territoires relative à la finalisation des DPE dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments.

je me réjouis que le Gouvernement s'engage sur la fiabilité de ce dernier, et j'ai trouvé Mme la rapporteur quelque peu défaitiste dans sa présentation du DPE.

au 1 janvier 2020 et qu'on ne dispose pas d'une étude d'impact permettant d'évaluer avec précision les conséquences de cette opposabilité en termes de contentieux pour les entreprises entreprises et en matière de vente et de location de logements. En outre, selon les professionnels du bâtiment, les consommations réelles des bâtiments dépendent très directement des conditions d'usage et de la température effective de chauffage. Les consommations qui sont estimées dans un DPE ne peuvent donc absolument pas être garanties.

est ainsi libellé : La parole est à M. Fabien Gay. La transition énergétique et écologique est l'une des questions essentielles de notre temps. Nous voulons même inscrire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution, fut-elle déjà partie prenante de ce texte depuis le vote de la Charte de l'environnement. Toujours est-il que cette transition ne peut continuer Toujours est-il que cette transition ne peut continuer de n'être qu'une sorte de catalogue de bonnes intentions parfaitement louables, assorti d'une série de normes à respecter, ainsi que nous le voyons un peu avec le présent chapitre. Réduire les Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments est une forme de nécessité, l'habitat étant une source non négligeable d'émission de gaz à effet de serre. Il nous semble cependant qu'il convient de ne pas nier qu'une bonne partie des Françaises et des Français, issus de familles modestes, qu'ils soient locataires ou non, sont confrontés à de telles difficultés financières qu'il importe de leur donner les moyens de participer au grand élan collectif de préservation de l'environnement. secteur du logement social, il n'est pas très compliqué pour un bailleur de mettre en oeuvre une opération de remise à niveau écologique, les choses sont plus complexes pour les propriétaires isolés ou dans les copropriétés. Pour être précis, compte tenu des processus de financement échelonné de ce type d'opérations, il arrive un moment où il y a, au coeur de l'opération, une insuffisance de trésorerie qu'il conviendrait, nous semble-t-il, d'éviter, ne serait-ce que pour permettre à l'ensemble des immeubles destinés à connaître une opération d'amélioration des performances thermiques d'en être l'objet et sans mettre en cause l'engagement du ou des propriétaires de l'immeuble. Nous proposons donc que soit mis en place un dispositif de prêt sans intérêt, destiné à assurer la fluidité de l'opération sur le plan financier, à éviter l'arrêt brutal de celle-ci et à permettre, de fait, sa réalisation. Ce prêt serait, dans son esprit, assez proche de ce qui a été mis en place dans le cadre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, afin de garantir une meilleure trésorerie aux entreprises bénéficiaires. Il pourrait, par exemple, être versé directement au syndicat de copropriétaires, aux fins d'une juste allocation des ressources ainsi mobilisées.

prématurée, une expérimentation de la future réglementation thermique et environnementale pour les constructions nouvelles étant en cours. Celle-ci a, en effet, été lancée à la demande des pouvoirs publics et en concertation avec les acteurs du secteur pour répondre aux objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L'intégration du critère carbone dans la future réglementation fait consensus. En revanche, les exigences de la future réglementation environnementale doivent rester cohérentes avec le référentiel en cours d'expérimentation, qui intègre des critères couvrant largement la performance environnementale. Aucune exigence nouvelle en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments, de recours à des matériaux renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, ou encore de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments ne paraît donc justifiée.

sont non conformes ou non fonctionnelles, ce qui fait de cette problématique un enjeu de santé publique, en plus d'être un enjeu en termes d'efficacité énergétique. Le ministère mène des travaux sur le sujet et la réglementation RT 2012

... À ce jour, aucun contrôle obligatoire à réception de ces installations de ventilation n'est prévu par la réglementation. C'est pourquoi cet amendement vise simplement à remédier à cette situation, en instituant, dans la loi, la définition par décret d'un contrôle des systèmes de ventilation, comme il en existe déjà un pour ce qui concerne la vérification de la valeur de la perméabilité à l'air du bâti au sein de la réglementation thermique, étant rappelé que l'objectif n'est pas d'ajouter pas d'ajouter des dépenses supplémentaires. Les modalités de ce contrôle peuvent être diverses pour éviter des coûts supplémentaires.

en introduisant la prise en compte de l'empreinte carbone de ceux-ci sur l'ensemble du cycle de vie. Il tend à encourager le recours aux matériaux capables de stocker du carbone de l'atmosphère, tels que les matériaux issus des ressources renouvelables. Cet amendement vise à apporter une modification rédactionnelle, ainsi que des précisions, notamment quant à l'évaluation du stockage de carbone, qui doit être réalisée tout au long du cycle de vie du bâtiment et non pas uniquement lors de la phase de construction ou de démolition. Quel

L'amendement n° 114 rectifié tend à cibler explicitement des exigences sur les systèmes de ventilation, ce qui conduirait à une interprétation de la loi

a vocation à rassembler les informations numérisées portant sur l'entretien du bâtiment, ses caractéristiques, ainsi qu'une mémoire des travaux réalisés, notamment à des fins d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Or ce carnet reprend essentiellement des données d'ores et déjà requises par différentes réglementations qui n'ont qu'une valeur informative. Il peut cependant être mis en oeuvre volontairement par les personnes concernées- les propriétaires ou les gestionnaires d'immeubles -sans qu'aucune intervention du législateur soit requise. Compte tenu de l'imprécision existante, la mesure proposée, en renvoyant le soin au pouvoir réglementaire de fixer les modalités d'application qui recouvrent en réalité la définition de l'objet du carnet numérique déjà consacré par l'actuel article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation,

intéressant à valeur informative.

L'article 55 a pour objet de préciser les fonctions de ce document et d'élargir son champ d'application pour faciliter sa mise en oeuvre effective. La commission a décidé, de manière difficilement compréhensible, de sortir le logement social du champ d'application du carnet. De plus, dans son rapport, elle ne motive même pas cette exception, précisant que le droit en vigueur exclut le logement social du dispositif,

cet amendement, il s'agit bel et bien de créer une cohérence entre les grands dispositifs territoriaux à l'échelle des intercommunalités, le PLH et le PCAET.

qui coordonneraient l'ensemble des acteurs et des actions existantes, et orienteraient davantage de particuliers souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique vers le service public de la performance énergétique de l'habitat. Cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné.

Cet amendement a donc pour objet de lancer un appel à projets pour désigner plusieurs territoires pilotes dans lesquels serait expérimentée une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Cette stratégie viserait à coordonner les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique, et à massifier les opérations de rénovation.

une ou plusieurs personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine une peine de confiscation générale de leur patrimoine, comme c'est le cas en matière de blanchiment. La confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l'absence de tout lien avec l'infraction, ainsi que sur tous les biens

de 75 000 euros à 375 000 euros. En effet, le nombre de condamnations de bailleurs exposant leurs locataires à des risques pour leur sécurité et leur santé est certes en hausse, mais reste faible au regard de la réalité du phénomène des marchands de sommeil. L'expérience montre que la lutte contre l'habitat indigne est particulièrement difficile à mettre en oeuvre. Les procédures sont complexes à engager et souvent mal appréhendées. Elles sont longues, puisqu'elles parfois davantage, et les résultats sont rarement à la hauteur des attentes, puisqu'ils n'atteignent pas toujours leur cible. Ces situations mal vécues par les habitants

en augmentant le montant de l'amende pour le délit de divulgation de l'identité d'un témoin, portant de 75 000 à 375 000 euros, ce qui est effectivement considérable,

a en réalité une portée tout à fait générale et aurait vocation à s'appliquer à toutes les procédures pénales. Le fait de révéler l'identité d'un témoin ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est déjà puni dans les textes de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Indépendamment de cet aspect, l'augmentation dans de très fortes proportions de l'amende pose un problème au regard du principe constitutionnel

qui permettent le repérage jusqu'à ceux qui ont un caractère incitatif ou coercitif, et renforcer la capacité d'action des pouvoirs publics. Notre amendement a pour objet de permettre aux collectivités locales, sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil, de bénéficier de la confiscation de ces biens à l'issue des procédures pénales. fois la peine complémentaire de confiscation de l'usufruit ou de confiscation des biens prononcée, elle pourra s'exercer au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui permettra à celles-ci de réaffecter l'usage de ces biens au logement social. Quel est

toutes les collectivités locales le souhaitent. Il se trouve en effet que la gestion des biens confisqués constitue une mission particulièrement technique et complexe. C'est pourquoi l'État a créé une agence dédiée. Les biens confisqués aux marchands de sommeil sont souvent en très mauvais état. Confier leur gestion aux collectivités territoriales nécessiterait

Monsieur le ministre,

des biens des marchands de sommeil qui auront été condamnés de manière définitive. À cet effet, nous avons prévu que la confiscation se fasse au profit

en l'étendant à l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, ou à la direction d'une entreprise commerciale ou industrielle. Globalement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons que je viens d'exposer. On continuera le travail entamé, mais je crois que les dispositions

vis-à-vis de son bailleur pendant la période intermédiaire entre l'arrêté de police générale pris en urgence, à la suite d'un incendie, par exemple, et la prise d'un arrêté de police spéciale relevant, par exemple, du péril ordinaire. Cette période intermédiaire suppose un certain temps d'instruction. La suspension du loyer permet de lever une difficulté subie par le locataire, à savoir le paiement du loyer d'un logement qu'il ne peut plus occuper. Cette précision permet ainsi de protéger les occupants des logements concernés par une mesure de police générale visant à les mettre à l'abri en raison d'un danger grave et immédiat. Quel est l'avis de la commission elle y sera défavorable. L'idée est intéressante et assurément à creuser, mais sa mise en oeuvre, en l'état, ne nous semble pas satisfaisante. En effet, dans le cadre de la police spéciale de l'insalubrité, le loyer et la durée du bail peuvent être suspendus, mais uniquement, dans

comme cela existe pour le blanchiment, et ce au-delà des seuls biens qui ont servi à commettre l'infraction. Quel

de prononcer la confiscation partielle ou générale du patrimoine des marchands de sommeil condamnés pour un hébergement contraire à la dignité humaine. Cette confiscation porte sur tout le patrimoine, et non sur le bien qui a servi à l'infraction, telle que nous l'avons systématisée.

puisse avoir omis de préciser qu'il s'agissait d'une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens, et non de la totalité des biens. Il appartiendra au juge de déterminer,

: La parole est à Mme Martine Berthet. La division d'un immeuble existant en vue de créer plusieurs locaux à usage d'habitation sans autorisation d'urbanisme est permise afin de densifier le foncier bâti, donc de limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et fait naître un risque sérieux d'insalubrité. Le code de la construction et de l'habitation prévoit qu'une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer. Le présent amendement vise à supprimer cette condition, permettant ainsi à l'ensemble des EPCI compétents en matière d'habitat ou, à défaut, à l'ensemble des conseils municipaux, sans condition, d'instaurer une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant.

quasi-automaticité du prononcé des peines complémentaires, comme celle de confiscation d'un bien ayant servi à commettre l'infraction. Afin d'assurer une meilleure lisibilité de ces mesures, l'amendement de réécriture

qui était source de réduction de la rentabilité des placements financiers concernés et, par voie de conséquence, de mise en réserve de moyens d'amélioration ultérieure du confort des logements concernés. Il est toutefois intéressant que, après quatre décennies d'application de la loi de 1948 et d'expansion du logement locatif social, au travers de la construction de nombreuses cités HLM, sous des conditions de financement particulièrement favorables, nous soyons passés à un renchérissement des opérations de logement social, avec le dispositif des prêts locatifs aidés, et à l'alourdissement des loyers, sous forme de « dérapage contrôlé l'expression n'est pas de moi -, avec le conventionnement et la montée en puissance de l'accession à la propriété. Mais cela ne suffisait pas encore et, plutôt que de répondre aux besoins de logements en partant de la situation de la demande, on a uniquement développé une politique de l'offre. Vous en connaissez les résultats : hausse continue des loyers et émergence des tensions. Le décalage croissant entre l'offre et la demande a été encouragé, comme nous l'avons déjà souligné. Il s'est également matérialisé dans la réémergence de l'habitat sans confort, que l'on croyait disparu au terme des opérations de restauration urbaine des centres historiques de nos grandes villes des années soixante et soixante-dix. La lutte contre l'habitat indigne et insalubre, dont la constitution a notamment été favorisée par les congés

Cette action exemplaire contre l'habitat indigne et insalubre se mène notamment au travers de structures de coopération interinstitutionnelle : je veux parler des pôles départementaux

vous proposez de reconnaître, au niveau législatif, l'existence des pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne, dont nous nous accordons tous à reconnaître qu'ils sont des outils indispensables au bon fonctionnement de cette politique publique.

figurer dans la loi une description formelle de ces instances de coordination, qui relèvent, en fait, de l'organisation interne tant de l'État que des collectivités territoriales.

paraît opportun de clarifier la législation sur les critères de superficie permettant d'apprécier l'état de suroccupation, dans le sens des dispositions fixées par le législateur et de l'amélioration des conditions de vie effectives des locataires.

contourner par les marchands de sommeil. De plus, dans la mesure où le décret de 2002 autorise une surface de 9 mètres carrés, de nombreux logements- je pense, par exemple, aux chambres de service -pourraient être qualifiés d'insalubres du jour au lendemain, en raison de leur surface inférieure à 14 mètres carrés.

le relogement est assuré par une personne publique, un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif, le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble insalubre lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement égale à un an du loyer prévisionnel. Or cette somme ne suffit pas à faciliter les relogements. Il est donc proposé d'augmenter l'indemnité exigible auprès du bailleur indélicat ou du marchand de sommeil à l'équivalent de trois ans de loyer. Quel

le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande. Notre amendement vise à préciser que son rapport doit être transmis à l'autorité compétente et aux occupants concernés dans les trois mois suivant le constat. Quel est

en matière d'aide sociale et de santé délègue aux collectivités territoriales les règles générales d'hygiène, un règlement sanitaire départemental type, dit RSDT,

Or les procédures en matière d'insalubrité dans l'habitat ont considérablement évolué, sans articulation avec le RSDT. La loi du 6 janvier 1986 suscitée

Cette carence a pour conséquence un défaut d'articulation entre le règlement sanitaire départemental, les procédures d'insalubrité et les dispositions qui protègent les victimes des marchands de sommeil. On observe fréquemment que les enquêtes conduites par les agents des services communaux ou intercommunaux de l'hygiène ne sont pas transmises aux services de santé de l'État et se bornent à transmettre une injonction, voire une amende, laquelle se monte au maximum à 450 euros. Cette situation laisse les locataires aux mains de leur marchand de sommeil. Il est cohérent de fixer un délai au Gouvernement pour publier ce décret attendu depuis

? Cet amendement a pour objet de contraindre l'État à adopter un décret relatif à la salubrité des habitations, laquelle est traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental.

à compter de la promulgation de la loi pour la publication du décret en Conseil d'État destiné à remplacer les règlements sanitaires départementaux en ce qui concerne la salubrité des habitations. Comme vous l'avez rappelé, ce décret en Conseil d'État était prévu par la loi du 6 janvier 1986, mais n'a jamais été publié pour le volet concernant la salubrité des habitations. cela montre que, malgré toutes ses vertus, la V République a encore quelques problèmes

Il permet aux représentants de l'État à Mayotte et en Guyane de procéder à l'évacuation et à la démolition des bidonvilles, dans des conditions d'efficacité renforcées, comme le résume le rapport.

en la forme des référés. Cette procédure dérogatoire est, à notre sens, inacceptable. Le Sénat s'honorerait à la supprimer.

Finalement, avec l'article 57, ces infortunés construiront ailleurs, sans aucune garantie supplémentaire de légalité et de salubrité, des habitations que le préfet s'empressera sûrement de démanteler, pour les mêmes raisons et selon la même procédure.

Au lieu de financer des démantèlements, finançons plutôt l'amélioration massive et progressive de l'habitat et de son environnement- toitures, dallage, latrines, construction de ruelles

Mayotte pour une mise en oeuvre accélérée du plan Logement d'abord. Si cette situation est source d'importants troubles à l'ordre public, comme le souligne le Gouvernement dans son exposé des motifs, n'oublions pas qu'elle est aussi source de colère et de révolte chez les populations

L'importance du nombre de logements dits informels et leur concentration dans des bidonvilles comme Kawéni à Mamoudzou ou Caro-Bolé à Koungou exigent une réponse appropriée. Les populations vivant dans ces quartiers, souvent étrangères en situation régulière ou de clandestinité, sont en effet exposées à des risques naturels élevés et à des conditions sanitaires propices au développement d'épidémies. Face à cette situation, la ministre des outre-mer estime que, à Mayotte comme en Guyane, le retard en construction de logements n'est pas rattrapable, non du fait d'insuffisances budgétaires, mais parce que les nécessaires ressources, notamment en main-d'oeuvre qualifiée, sont peu nombreuses. Néanmoins, le Gouvernement entend faire passer le nombre de constructions annuelles de 300 à 800 logements. Le projet de loi donne au préfet la possibilité d'expulser les occupants d'habitats

Cette solution n'offre aucune alternative aux résidents en termes de relogement, si ce n'est une proposition d'hébergement d'urgence pour une nuit seulement, alors que leur habitat peut avoir été édifié depuis plus d'une décennie.

monsieur le ministre,

que nous avons apporté des garanties relatives à l'hébergement, au relogement et à la bonne information des personnes évacuées.

à compléter les dispositions existantes pour permettre aux préfets de Mayotte et de Guyane de procéder aux démolitions de locaux et d'installations sans qu'il soit nécessaire d'obtenir préalablement une ordonnance du juge et un avis du CODERST. Pour garantir les droits des occupants, ce même article prévoit un délai minimal d'un mois pour procéder à l'évacuation, la possibilité de saisir le juge en référé et l'obligation du préfet

ministre. Monsieur le sénateur, vous avez rappelé, à juste titre, que cette situation ne remonte pas au mois de juin 2017. Je ne pense pas que M. Iacovelli dise autre chose.

en Guyane, plusieurs opérations NPNRU sont en train d'être lancées sur le secteur de l'habitat informel.

chantage, expulsion illégale ... Cette loi du silence organisé nuit à l'efficacité de la lutte contre l'habitat indigne. Cet amendement vise à préciser, dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance, la protection et les droits des habitants de locaux indignes. Quel

de la qualité sanitaire des bâtiments et l'article 50 exige du propriétaire mettant en location son bien qu'il soit exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites.

Le deuxième tend à rétablir une disposition qui avait été supprimée lors de l'examen de la loi Macron au motif que ce n'est pas le transport de la mérule qui engendre son développement. Je ne vois pas pourquoi, trois ans après, cela aurait changé ... Le troisième permet au maire d'enjoindre à l'occupant de procéder, dans les six mois, à la recherche de mérules et aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

au propriétaire et au syndicat des copropriétaires de procéder dans les six mois à la recherche de mérules ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.

la notion de violation de domicile est d'ores et déjà lourdement sanctionnée et les juges sont peu laxistes sur la question. La distinction entre un bien occupé et un bien vacant est essentielle au respect de la proportionnalité des peines et de la nécessité de la loi pénale. Certes, un propriétaire doit pouvoir récupérer son bien vacant, mais cela ne peut pas se faire hors des règles applicables. L'impact n'est pas le même selon qu'il s'agit ou non d'une occupation de la résidence principale. La procédure express prévue par la loi DALO pour l'occupation du logement principal a été conçue pour être dérogatoire et n'a pas à se retrouver dans le droit commun. Enfin, le préfet n'a pas à se substituer aux juges et à rendre justice, hormis dans les cas d'urgence d'occupation de la résidence principale, puisque le propriétaire se retrouve alors à la rue. Le caractère opportuniste de ces amendements récurrents ne doit pas nous faire oublier le problème réel du mal-logement. Les logements vacants représentent, nous l'avons déjà dit au cours de nos débats, plus de 8 % du parc de logements en France, soit près de 3 millions de logements. Or les occupants de logements vacants peuvent être des familles en situation précaire avec des enfants en bas âge. Les expulsions doivent en tenir compte, d'où la nécessité de la décision d'un juge, qui analyse les intérêts des deux parties. C'est également la raison de certains délais qui peuvent parfois être accordés lorsqu'il ne s'agit pas du domicile du propriétaire.

qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. La

Cela ne revient pas, comme vous avez semblé le dire, à réduire le champ des biens protégés, mais au contraire à l'élargir, afin d'être beaucoup plus performant dans la lutte contre les squats, qui constituent un véritable fléau.

Afin de lutter efficacement contre cette situation, je veux rappeler le travail de notre collègue Catherine Procaccia, qui avait fait adopter un amendement à la loi du 5 mars 2007, dite loi DALO, punissant l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui par le biais de l'article 226-4 du code pénal, évoqué tout à l'heure par M. le secrétaire d'État. Néanmoins, malgré cette heureuse avancée, notre droit pénal demeure insuffisant pour réprimer efficacement cette infraction. En effet, la notion de flagrant délit qui permet une expulsion rapide des squatters est difficile à caractériser. Au-delà de 48 heures - c'est un délai très court -suivant l'intrusion, le flagrant délit n'est plus caractérisé et la police ne peut donc plus procéder à l'expulsion immédiate. Il est alors nécessaire d'obtenir une décision judiciaire au terme d'une longue et laborieuse procédure. Le délai de 48 heures nous semble donc trop court pour permettre aux propriétaires d'actionner une procédure d'expulsion immédiate auprès des forces de police.

contrainte d'émettre un avis défavorable. Il ne nous a pas paru opportun d'introduire dans cet article général, qui concerne l'ensemble des crimes et délits, un délai spécifique pour l'infraction de violation de domicile. Plus globalement, il n'est pas utile d'apporter une première dérogation au principe de l'absence de fixation de durée fixe pour constater la flagrance d'une infraction, quelle qu'elle soit. De plus, limiter la durée de la flagrance à 96 heures à compter de la commission de l'infraction peut s'avérer contraire à l'intérêt de la victime. Si celle-ci est absente pour une durée supérieure - hospitalisation, vacances, voyage à l'étranger - et que, pendant son absence, le maintien du squatteur dans les lieux se poursuit, à son retour,

dont celle du maintien dans le domicile d'autrui, qui présente la particularité d'être une infraction continue et non une infraction instantanée, comme l'est l'introduction dans le domicile d'autrui. C'est cette particularité qui permet aux forces de l'ordre, tout au long de l'occupation - je dis bien tout au long de l'occupation - d'intervenir et d'interpeller les squatteurs, quel que soit le délai écoulé. On n'arrive pas à se faire entendre sur ce point ! Qu'on me dise que la difficulté est liée à l'exécution, c'est-à-dire à l'intervention des forces de l'ordre, je peux l'entendre l'entendre ! Mais les dispositions légales ne sont pas en cause. On peut agir après introduction dans le domicile plus de 48 heures après l'infraction, puisque les services de police peuvent agir en flagrance pendant toute la durée de l'occupation.

existant, le flagrant délit pouvant être constaté non seulement 96 heures après le début de la commission de l'infraction, mais aussi durant toute la durée de l'infraction.

On ne peut pas prévoir de dérogation en introduisant un délai de flagrance particulier pour un délit spécifique, sauf à faire perdre à la procédure pénale son caractère d'unicité, ce qui n'est pas, à l'heure de la simplification, le souhait du Gouvernement. le souhait du Gouvernement. J'ai expliqué et réexpliqué cela non seulement lors de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale, mais aussi dans le cadre d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par le groupe